Mes chers collègues, au regard de notre ordre du jour, et afin d'éviter tout risque de report de mission, j'invite chacun et chacune d'entre vous à la concision et au respect du temps de parole. La parole

madame la ministre, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances », qui porte les politiques publiques de solidarité et de cohésion sociale de l'État en faveur des personnes les plus fragiles,

Cette augmentation est principalement due au dynamisme des dépenses d'intervention, qui représentent 93 % des crédits de la mission, mais s'explique également par les revalorisations dites « exceptionnelles » de la prime d'activité et de l'allocation aux adultes handicapés. Il y a ainsi un effort budgétaire d'ensemble de la part du Gouvernement, que nous reconnaissons, mais qui doit cependant être nuancé par l'existence d'un certain nombre de mesures de paramètre, des mesures dont l'impact sur les bénéficiaires ne semble, d'ailleurs, pas vraiment maîtrisé par le Gouvernement, ce qui est quelque peu inquiétant. Derrière la communication gouvernementale et les revalorisations annoncées, la réalité des crédits de la mission atteste, en effet, de la mise en oeuvre d'un certain nombre de réformes de paramètre, qui viennent minorer, voire neutraliser dans certains cas, les revalorisations annoncées, le Gouvernement ayant choisi de faire sien le célèbre adage « donner d'une main pour mieux reprendre de l'autre » ... En effet, parallèlement aux revalorisations annoncées, différentes mesures sont prévues par le projet de loi de finances pour 2019, ou ont déjà été mises en oeuvre par la loi de finances pour 2018. Concernant tout d'abord la prime d'activité, il s'agit de la baisse de l'abattement portant sur les revenus d'activité pris en compte dans le calcul de la prime- de 62 % à 61 %-, intervenue par un décret d'octobre dernier. Ainsi, d'après des simulations effectuées, sur les 20 euros de revalorisation forfaitaire annoncés, une personne au SMIC et sans enfant bénéficierait d'un gain de seulement 8 euros Autre réforme paramétrique, l'exclusion pour les « nouveaux entrants » du bénéfice de la prime d'activité : les bénéficiaires de rentes accidents du travail décidé la suppression de la revalorisation annuelle du 1 avril pour 2019 et 2020 de la prime et de son bonus, indexées jusque-là sur l'inflation. De même, pour l'allocation aux adultes handicapés, l'AAH, sont prévues ou déjà mises en oeuvre les réformes de paramètre suivantes.

Outre le fond de ces mesures, c'est surtout la méthode du Gouvernement qui est quelque peu critiquable, madame la ministre. Le Gouvernement a su abondamment communiquer sur les coups de pouce, en oubliant d'évoquer ces nombreux coups de ciseaux, qui seront autant de mauvaises surprises pour les bénéficiaires,

et notamment les simulations réalisées par le Gouvernement, pour connaître le réel impact de toutes ces mesures de restriction budgétaire sur les bénéficiaires. Nous nous sommes essayés à l'exercice et avons obtenu des ordres de grandeur, mais nous aimerions avoir des chiffres plus Malgré ces insuffisances, que je regrette, la commission des finances a décidé d'adopter ces crédits, mais également de voter un amendement visant à maintenir, conformément au droit existant, le complément de ressources à l'allocation aux adultes handicapés. La parole est

la mise en oeuvre du budget de la mission, pour 2019, est entourée d'un certain nombre d'incertitudes. Elles concernent notamment le financement des mineurs non accompagnés. L'aide exceptionnelle aux départements s'agissant de la prise en charge partielle des dépenses d'aide sociale à l'enfance est certes reconduite, mais l'incertitude demeure sur son montant. Il semblerait que le niveau des dépenses prises en charge par l'État diminue, passant de 30 % à 15 %. Toutefois, malgré nos demandes, le Gouvernement n'a malheureusement pas été en mesure de nous le confirmer, ce qui est regrettable, puisqu'une enveloppe a bien été budgétée pour 2019. Nous souhaiterions, madame la ministre, avoir, sur cette question, des éléments de réponse de votre part. Par ailleurs, sur ce sujet qui relève, à notre sens, de la politique nationale d'immigration, nous estimons que l'État doit prendre ses responsabilités, d'une part, en assumant les dépenses d'évaluation et de mise à l'abri, et, d'autre part, en augmentant l'aide versée aux départements pour les dépenses d'aide sociale à l'enfance. Outre cette question des MNA, il est un autre sujet dont l'exécution nous semble entourée d'incertitudes : il s'agit du plan Pauvreté. Nous ne pouvons que saluer les objectifs de cette stratégie et le travail mené par le délégué interministériel, que nous avons reçu en audition. Néanmoins, la majorité des crédits inscrits au titre de la mission reposent sur une contractualisation avec les départements. La mise en oeuvre de ce plan semble ainsi, en l'état actuel des choses, compromise au vu de la situation financière des départements. Un autre sujet était entouré d'incertitudes, et le Gouvernement est finalement intervenu en cours de discussion à l'Assemblée nationale : la suppression de la prise en compte, en tant que revenus professionnels, des rentes AT-MP et des pensions d'invalidité dans le calcul du droit à la prime d'activité. Cette mesure avait été adoptée en loi de finances initiale pour 2018, contre l'avis du Sénat, pour une application au 1 janvier 2018. Elle fut appliquée temporairement, et avec retard, au 1 juin 2018, mais le Gouvernement a finalement « fait machine arrière », suspendant l'application de la mesure au vu de ses conséquences dommageables sur les bénéficiaires, conséquences que l'on avait pourtant pointées lors de l'examen de la dernière loi de finances. Des pertes ont ainsi été constatées chez les bénéficiaires- majoritairement, des familles monoparentales -s'échelonnant de 60 à 200 euros par mois. On ne peut que regretter, madame la ministre, madame la secrétaire d'État, la mise en oeuvre chaotique de cette mesure, qui n'a fait l'objet d'aucune publicité auprès des bénéficiaires, ni s'agissant de la suppression du droit ni ensuite s'agissant du versement du rappel. Nous reviendrons, lors de l'examen des amendements, sur l'article que vous avez ajouté, par voie d'amendement, à l'Assemblée nationale. Enfin, le dernier financement entouré d'incertitudes que je souhaitais aborder ici dépasse le cadre strictement national. Il s'agit du financement de l'aide alimentaire par le biais du Fonds européen d'aide aux plus démunis, dont nous avons montré le caractère essentiel dans un récent travail de contrôle sur le sujet. Nous souhaiterions, à l'heure où les négociations européennes débutent, que le Président de la République et le Gouvernement s'engagent clairement pour la pérennisation de ce fonds. Enfin, je terminerai mon intervention par un mot sur les deux autres programmes de la mission. S'agissant du programme 137 relatif à l'égalité entre les femmes et les hommes, ses crédits sont stables à l'euro près, mais masquent des situations contrastées, notamment la diminution des crédits liés à la lutte contre la prostitution, portée par la loi du 13 avril 2016. Bien que la diminution soit moins importante que l'année dernière, nous tenions à rappeler que le maintien de financements aux associations est essentiel, puisque d'elles dépend la mise en oeuvre de cette loi et des parcours d'accompagnement de sortie de la prostitution. Enfin, s'agissant du programme 124- il porte l'ensemble des crédits de soutien des politiques des ministères sociaux et la contribution de l'État au fonctionnement des agences régionales de santé -, ses crédits diminuent de près de 2,5 %. Les ministères sociaux faisant partie des ministères non prioritaires, ils sont ainsi touchés significativement, depuis plusieurs années, par des mesures d'économie budgétaire. Il semble néanmoins que le processus de rationalisation des moyens atteigne aujourd'hui ses limites. Nous serons ainsi attentifs, mesdames les ministres, au maintien d'un niveau satisfaisant des crédits en cohérence avec le bon fonctionnement de ces ministères. Ainsi, pour ces différentes raisons, j'avais, personnellement, émis un avis défavorable à l'adoption des crédits de cette mission. La commission des finances a finalement décidé de les adopter. La parole est à M.

madame la ministre, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, je suis rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales sur les crédits de la mission depuis quatre ans. Bien que cette période ait vu une augmentation régulière de ces crédits, je constate une évolution moins solidariste des politiques publiques qu'elle finance. La prime d'activité nous en fournit depuis deux ans l'illustration. Voilà une prestation sociale dont le succès, certes, ne se dément pas, mais dont l'objectif repose sur une ambiguïté : minimum social ou incitation financière au retour à l'emploi La réduction de la pauvreté est un objectif évidemment louable, mais encore faut-il qu'il soit mesuré à partir de principes fermement établis, et pas simplement à l'aune de dépenses budgétaires reconduites, année après année, sans que le cap soit clairement défini. La prime d'activité repose sur deux composantes : l'une familialisée et l'autre individuelle. Selon l'arbitrage, un effort concentré sur la première contribuera à l'augmentation du niveau de vie des ménages les plus pauvres, alors que la seconde touchera davantage l'incitation financière au retour à l'emploi. Par les mesures contenues dans le présent projet de loi de finances, le Gouvernement privilégie ce dernier aspect, limitant ainsi le soutien aux revenus les plus modestes. Le programme dispersé de la stratégie pluriannuelle de prévention et de lutte contre la pauvreté, qui sera majoritairement orienté vers l'insertion dans l'activité, promet, certes, de belles réussites, mais laisse présager d'inquiétantes lacunes ... Tandis que les efforts porteront sur les « moins pauvres des plus pauvres », qu'en sera-t-il des autres ? Les mesures qui les visent directement sont d'une ambition moindre et, surtout, ne paraissent pas encore parfaitement abouties : crèches à vocation sociale et « petit-déjeuner pour tous » sont dénoncés par certaines associations comme inopérants. sont susceptibles d'en faire le meilleur usage, on attribue les revenus de remplacement réévalués ; aux autres, on réserve les prestations en nature : curieuse partition ... Un autre sujet de la mission doit être évoqué : la réforme de l'allocation aux adultes handicapés. La revalorisation de son montant, qui passera à 900 euros d'ici au 1 novembre 2019, est une excellente nouvelle. Je tiens néanmoins à rappeler mon attachement au caractère spécifique de l'AAH et au danger qu'il y aurait à calquer sur cette prestation, créée pour des personnes en situation d'inadaptation durable à l'emploi, les critères généraux des autres minima sociaux, conçus, eux, pour inciter à la reprise d'une activité. de rapprochement de l'AAH et du RSA, qu'illustre notamment la fusion des compléments de ressources, présente selon moi le danger de la perte d'une spécificité qu'il faut maintenir. Enfin, la commission des affaires sociales a adopté un amendement visant à créer, sans modification de crédits, un nouveau programme budgétaire spécifique à l'évaluation et à l'hébergement d'urgence des mineurs non accompagnés,

mes chers collègues, malgré son intitulé, la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances » est loin d'épuiser à elle seule les moyens que la Nation consacre à la solidarité envers nos concitoyens en difficulté et à la réduction des inégalités. sécurité sociale pour 2019 consacre cette année 500 milliards d'euros au financement de la protection sociale, qui est au coeur de notre système solidaire. La mission « Travail et emploi » est l'un des autres vecteurs de la solidarité, avec des crédits majoritairement consacrés à l'insertion dans l'emploi. Je pourrais aussi convoquer le budget de l'éducation nationale de l'enseignement supérieur, dont l'objet même est d'offrir à nos futurs concitoyens les outils indispensables à l'égalité des chances que sont le savoir et les compétences. Tant par les prélèvements que par les prestations, le système socio-fiscal français est un puissant moteur de réduction des inégalités, qui concrétise au quotidien le troisième terme de la devise de la République. Aux côtés de l'État régalien, celui de la défense, de la police et de la justice, il y a donc bien un État social, auquel est consacré près d'un tiers de notre richesse nationale. Le modèle social français divise ainsi par quatre les écarts de revenus entre les 10 % les plus riches et les 10 % les plus pauvres. Cet effort ne s'est pas démenti pendant la crise, notre pays ayant fait le choix de l'augmentation des impôts, mais aussi des déficits pour garantir ce modèle, même s'il l'écornait quelque peu au passage dans son soutien aux familles, la baisse des prestations ayant suivi de peu la baisse du quotient familial. Les Français semblaient s'accommoder d'un haut degré de prélèvements pour garantir cette spécificité qui semblait placée au coeur de notre identité. Comment se fait-il, alors, que ce modèle semble craquer de toutes parts depuis quelques semaines, déchiré entre des injonctions contradictoires de « plus de solidarité » et de « moins d'impôt » Dans ces circonstances complexes où les passions se mêlent aux contradictions, on ne peut que faire preuve d'humilité dans la recherche d'explications. J'en tenterai cependant quelques-unes. La première, c'est que nous ne sommes pas sortis de la panne de croissance qui mine notre pays depuis trop d'années. La crise reste bien présente dans tous ses aspects crise économique, crise des finances publiques, crise sociale, elle est devenue une crise de confiance, dans l'avenir, dans les institutions, dans la possibilité pour les jeunes à vivre demain mieux que leurs parents. Dans les réponses apportées, les gouvernements successifs n'ont pas su éviter deux écueils majeurs. Le premier, c'est le piège du pouvoir d'achat, porté en étendard, alors que l'État est bien loin d'en maîtriser tous les paramètres, puisqu'il relève avant tout de la situation de l'emploi. Le second, c'est la tentation du meccano fiscal, certes irrésistible, parce qu'il entretient l'illusion de l'action, mais à la complexité si effroyable et aux résultats si limités qu'ils ne peuvent que semer le doute dans l'esprit de nos concitoyens quant à ses finalités ultimes. Quel besoin y avait-il ainsi d'emporter dans un même tourbillon la fiscalité du patrimoine, la contribution sociale généralisée, la taxe d'habitation et les cotisations sociales avec des effets et des calendriers différenciés ? Tout à fait ! Le résultat est en tout cas une incompréhension totale, un brouillage complet et une méfiance accrue. Derrière le débat, d'apparence technique, qui a émergé ces dernières semaines sur l'affectation de telle ou telle taxe à telle ou telle dépense au sein du budget de l'État, se profile un autre sujet d'ampleur, celui du consentement à l'impôt. La commission des affaires sociales s'est opposée, pour cette raison, aux modifications intervenues dans le financement de la sécurité sociale et de l'assurance-chômage. Les cotisations sociales ont un sens, celui de la contrepartie sous forme de prestation. Cette contrepartie que certains de nos concitoyens perdent de vue et ne perçoivent plus doit rester présente dans la sphère sociale. C'était le sens du rétablissement, par le Sénat, de la contribution salariale d'assurance chômage, dont nous considérons qu'elle n'est pas équivalente à une CSG devenue indifférenciée et sans doute trop élevée. Pour en venir plus précisément aux crédits de la mission qui nous occupe ce matin et qui traduit les premières orientations du plan de lutte contre la pauvreté, nous avons besoin de clarté, clarté sur les objectifs, clarté sur les bénéficiaires, clarté sur les résultats attendus.

en son temps devant notre commission, le débat entre soutien à la reprise d'activité et soutien au niveau de vie des familles n'est pas tranché et la lisibilité de cette prestation s'en ressent. Clarté sur les bénéficiaires des prestations, ensuite. Le retour en arrière sur la prise en compte des rentes AT-MP et des pensions d'invalidité en tant que revenus professionnels traduit, là encore, une certaine hésitation. Que voulons-nous faire de la prime d'activité ? Clarté sur les résultats attendus, enfin. Nous ne pourrons jamais garantir un revenu considéré comme satisfaisant par des revenus de transfert. Ils doivent néanmoins garantir une certaine dignité, en application du préambule de la Constitution de 1946, à ceux qui ne peuvent subvenir à leurs besoins par eux-mêmes. À tous les autres, la solidarité nationale doit garantir les moyens d'accéder à l'autonomie et d'exercer leur liberté en favorisant l'émancipation par la santé, par l'éducation et par le travail. Mes chers de finances pour 2019. Mes chers collègues, je vous rappelle que le temps de parole attribué à chaque groupe pour chaque discussion comprend le temps d'intervention générale et celui de l'explication de vote. Par ailleurs, le Gouvernement dispose au total de dix minutes pour intervenir.

La mission « Solidarité, insertion et égalité des chances » compte plusieurs mesures de soutien destinées à celles et ceux qui en ont le plus besoin. Elle s'inscrit totalement dans la volonté du Gouvernement de « faire plus pour ceux qui ont le moins

Parmi les mesures de solidarité de ce projet de loi de finances, la première vise à revaloriser dès avril prochain le montant de la prime d'activité de 30 euros au niveau du SMIC, par création d'un bonus. En quelques mois, c'est la deuxième augmentation, après la récente majoration d'octobre dernier. Ce bonus, croissant jusqu'à un SMIC, sera versé à chaque membre du foyer dont les revenus sont compris entre 0,5 et 1,2 SMIC. Il augmentera significativement le pouvoir d'achat des travailleurs et renforcera l'incitation à l'activité. De plus, une réorganisation des prestations complémentaires à l'allocation aux adultes handicapés est prévue pour rationaliser et mieux articuler le soutien aux personnes en situation de handicap. Lors de la lecture à l'Assemblée nationale, le Gouvernement a introduit par voie d'amendement l'article 83 ,qui met en place l'expérimentation d'une innovation dans le mode de délivrance du RSA en Guyane, à Mayotte et à Saint-Martin. Cette innovation consiste à distribuer le RSA un titre de paiement de type « carte prépayée Elle a pour objectif de permettre aux bénéficiaires de régler l'achat de biens et l'ensemble des services ce moyen de paiement. Cela prend pleinement en compte les difficultés des usagers au sein des territoires, notamment leur faible accès aux services bancaires à Mayotte. Enfin, je souhaite particulièrement insister sur un amendement déposé par notre groupe et qui prévoit des expérimentations de mise en libre distribution de protections périodiques dans différents lieux accueillant du public, et notamment les personnes les plus vulnérables. Sujet trop souvent éludé, la précarité liée aux règles est peu connue et peu traitée dans notre pays. indéniable que, faute de moyens, beaucoup de femmes dans notre pays se retrouvent dans l'impossibilité de se procurer des protections périodiques. Ainsi, lorsque l'on vit à la rue ou en centre d'hébergement, les règles représentent des moments particulièrement difficiles, humiliants, et impliquent de nombreuses complications pour de trop nombreuses femmes déjà vulnérables, parfois contraintes d'utiliser des morceaux de vêtements pour se protéger. Cette situation critique sur le plan sanitaire et sur

en cette période troublée que la violence sauvage utilise et que nous devons unanimement condamner, j'aurais vraiment aimé approuver les crédits de la mission « Solidarité, Hélas, ce gouvernement fait de la mystification auprès des plus vulnérables sa méthode. Derrière les grandes déclarations se cache tout de même un certain cynisme ; c'est intolérable ! Ainsi se nourrissent et s'accroissent un profond ressentiment dans la population et de la défiance à l'égard des élus. Christine Lagarde, que l'on ne peut soupçonner d'être une dangereuse gauchiste, accuse les élites d'être inconscientes de ce qui se passe. Ainsi, sur l'AAH, une augmentation, louable, des crédits de 5,1 % est annoncée. En réalité, cette mesure est accompagnée de la suppression pure et simple d'un droit essentiel pour les bénéficiaires, à savoir la garantie de ressources fixée à 998 euros, soit en dessous du seuil de pauvreté. Cette garantie vole en éclats avec la fusion, injustifiable et incompréhensible, du complément de ressources et de la majoration pour vie autonome. Elle entraînera, de surcroît, une perte de pouvoir d'achat de 75 à 179 euros pour les nombreuses personnes concernées. Les mesures contre les personnes en situation de handicap ne s'arrêtent pas là : diminution de 10 % de l'allocation aux adultes handicapées pour les couples de bénéficiaires, suppression de la prime d'activité aux travailleurs invalides-on leur doit un peu plus de reconnaissance et de respect augmentation des frais de tutelle après désengagement de l'État et désindexation de l'AAH. Sur la prime d'activité, on atteint des sommets en matière de supercherie.

Hélas, le bleu budgétaire au bas de la page 38 précise : « Le montant forfaitaire de la prime d'activité a fait l'objet d'une revalorisation exceptionnelle de 20 euros [ En parallèle, le coefficient de prise en compte des revenus est abaissé d'un point, passant de 62 % à 61 %. » Pourquoi ? fait 12 euros de moins sur les 20 euros promis à un salarié au SMIC. Excusez du peu ! Ainsi, l'augmentation se limitera à 8 euros- désindexés, soit moins de 7 euros en réalité -pour un SMIC, et à 14 euros pour un demi-SMIC, sachant que le périmètre aussi a changé. En dessous d'un demi-SMIC, pas de prime d'activité ! Les plus touchés sont, encore et toujours, les plus fragiles, notamment les femmes travaillant à temps partiel et, encore, les personnes en situation de handicap Comment peut-on agir ainsi : tromper et accabler ceux de nos concitoyens qui, accablés, le sont déjà, et ce pour quelques économies minimes, surtout au regard de l'argent distribué aux très riches ? et les femmes, c'est la grande cause du quinquennat, selon le Gouvernement. Eh bien, la grande cause n'échappe pas « à la poudre de perlimpinpin ». On refond en totalité les crédits, selon une géométrie quelque peu fantaisiste. Cela permet subtilement, pense-t-on, d'opérer des des coupes importantes. Ainsi assiste-t-on à une réduction de 500 000 euros pour l'accompagnement des personnes en situation de prostitution, et à une réduction de 400 000 euros du montant de l'allocation financière pour leur insertion sociale et professionnelle, soit une baisse de 20 % des crédits consacrés à cette politique indispensable de lutte contre la prostitution et d'insertion des êtres qui y étaient contraints. Votre proposition met en péril l'accompagnement social apporté par les associations agréées, qui font pourtant un travail remarquable sur nos territoires pour lutter contre contre les violences sexistes et sexuelles et accompagner les personnes qui en sont victimes. Le même sort est réservé aux actions en direction des personnes en difficulté. Le RSA n'est pas revalorisé

Tandis que l'Union européenne peine à reconduire ses aides, les difficultés risquent d'être considérables cet hiver. Par ailleurs, le Gouvernement divise par cinquante le montant de l'aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine, laquelle en 2017 à 200 000 euros en 2019. Cette action, décidée en 2016, s'inscrivait dans une politique globale et lucide de l'immigration, s'efforçant de limiter les sorties et de favoriser les retours. Mais c'était l'ancien monde La lutte contre la pauvreté, annoncée comme l'une des grandes priorités- mais qu'est-ce qui, dans les déclarations du Gouvernement, n'est pas prioritaire ? -, ressemble juste à un alibi pour tenter de se construire une image plus noble que celle qui lui colle désormais à la peau de gouvernement des très riches. Un montant de

Il est vrai que l'ambition est de faire participer les collectivités locales ... Comment croire encore à la parole du Gouvernement, qui, là encore, communique plus qu'il n'agit ? Enfin, les ministères sociaux sont parmi les plus touchés par les suppressions de postes. Après 287 en 2018, le Gouvernement supprime, cette année, 460 contradictoire avec les grandes et belles déclarations. Curieuse vision d'une politique sociale ambitieuse ! On compte de moins en moins de personnels pour la mettre en oeuvre. Un tel acharnement quasi clandestin contre les politiques sociales, contre la cohésion sociale, c'est la négation de nos traditions de solidarité. Or la solidarité est le fondement d'une société civilisée, selon la définition d'Edgar Morin. Elle devrait permettre à tout individu, quelles que soient ses différences, d'accéder à son maximum d'autonomie, de s'insérer dans les meilleures conditions, tant sur le plan social plan professionnel, de réussir sa vie sans être condamné par les conditions de sa naissance. Il est grand temps de changer d'orientation, d'engager des actions de lutte contre les inégalités plutôt qu'accroître celles-ci, de favoriser l'épanouissement de tous, d'offrir à chacun les conditions de sa réalisation, de rassembler la Nation derrière et autour d'un projet pour une société plus juste, plus douce, plus harmonieuse et plus solidaire.

C'est l'une des évolutions les plus favorables de ce projet de loi de finances. Cette mission s'articule autour de deux grands programmes, mettant en oeuvre la prime d'activité et l'allocation aux adultes handicapés, qui représentent, à elles deux, près de 90 % des crédits de la mission. Il est naturel de rappeler notre attachement à ces mécanismes de soutien, destinés aux personnes les plus vulnérables ou dans les situations les plus précaires, notamment les femmes qui élèvent seules des enfants, au nom de la solidarité nationale. Les crédits de la mission s'inscrivent donc logiquement dans la mise en place de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté présentée par le Président de la République le 13 septembre dernier.

qui traduit une double volonté : une politique d'incitation à la reprise d'activité et un soutien au pouvoir d'achat. Notons tout particulièrement l'amélioration apportée par l'adoption, à l'Assemblée nationale, d'un amendement du Gouvernement, qui aura pour effet, avec le versement de cette prime, d'augmenter le SMIC de 30 euros supplémentaires dès le mois d'avril 2019, puis de 20 euros les deux années suivantes, soit une hausse totale de 80 euros d'ici à 2021.

serait renforcé par une compensation plus juste des dépenses engagées, sur la base d'un forfait calculé par jeune évalué. Pour reprendre vos propos, cela « traduit la volonté du Gouvernement d'oeuvrer à l'avènement d'une nouvelle contractualisation entre l'État et les conseils départementaux dans la déclinaison des politiques sociales. Pour autant, notre rapporteur pour avis, M. Philippe Mouiller, a estimé que ce montant était très insuffisant par rapport aux besoins exprimés, qui sont difficiles à chiffrer, étant donné que leur évolution est assez rapide. Par conséquent, il nous proposera d'adopter un amendement visant à créer un programme budgétaire distinct au sein de la mission, exclusivement dédié à l'accueil des mineurs non accompagnés. Il souhaite ainsi envoyer un signal fort, en incitant l'État à assumer une mission dont les conseils départementaux ont toujours pensé qu'elle relevait de sa compétence exclusive, au titre de la politique migratoire. L'évaluation et l'hébergement d'urgence de jeunes migrants dont la minorité n'est pas encore établie doivent être pleinement conduits par l'État. Aux conseils départementaux revient l'accompagnement des jeunes reconnus mineurs au titre de l'aide sociale à l'enfance.

de cette mission témoigne de la volonté du Président de la République et du Gouvernement de renforcer la solidarité en direction des plus fragiles de nos concitoyens. Même si ce message

Madame la présidente, mesdames les ministres, mes chers collègues, le 13 septembre dernier, le Président de la République dévoilait sa stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté, dont l'ambition est de lutter contre les inégalités de destin et permettre une égalité des chances réelle. Cette priorité sociale affichée par le Gouvernement se traduit par une augmentation de près de 7 % des crédits de la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances

années. Si le Gouvernement explique vouloir concentrer ses efforts sur les personnes les plus en difficulté, cette désindexation risque de placer un certain nombre de foyers aux portes de la pauvreté. Sans remettre en cause la priorité donnée à la lutte contre la pauvreté, le sentiment de déclassement grandit au sein de la population, surtout de la population qui travaille, comme en témoigne le mouvement des gilets jaunes. Aussi, la présente mission budgétaire revêt un rôle plus que jamais central. Je m'attarderai sur les points les plus saillants de cette mission. Le programme 157, « Handicap et dépendance », regroupe les crédits consacrés à l'allocation aux adultes handicapés. Ceux-ci sont en hausse de 5,1 % par rapport à 2018, portant l'enveloppe à 11,9 milliards d'euros. Cette augmentation permet de concrétiser l'engagement du Président de la République en faveur de la revalorisation de l'AAH. L'aide à taux plein sera portée à 900 euros à la fin de l'année 2019. Cet investissement doit être salué à sa juste mesure. Cependant, quelques ajustements paramétriques contrastent avec l'engagement tenu. Pour n'en citer qu'un, l'alignement des règles de prise en compte des revenus d'un couple bénéficiant de l'AAH sur celles d'un couple touchant le RSA abaisse mécaniquement le plafond en deçà duquel un couple peut bénéficier de deux AAH à taux plein. Les associations de personnes handicapées alertent à juste titre. L'AAH est par nature différente du RSA et leurs objectifs divergent. C'est notre premier point de vigilance. vigilance. Le programme 304, « Inclusion sociale et protection des personnes », est le deuxième programme le plus important en termes de crédits mobilisés, avec 7,7 milliards d'euros demandés pour 2019, soit 1 milliard d'euros de plus qu'en 2018. Selon le Gouvernement, ce programme sera l'instrument majeur dans l'application de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté. L'un des outils mobilisés est la revalorisation de 20 euros, en 2019, du montant forfaitaire de la prime d'activité. succède à une première hausse du même montant, intervenue en 2018. D'ici à la fin du quinquennat, la revalorisation pour les bénéficiaires de la prime d'activité rémunérés au niveau du SMIC s'élèvera à 80 euros. Comme l'a souligné fort justement notre rapporteur pour avis, Philippe Mouiller, la concentration sur la prime d'activité des efforts de lutte contre la pauvreté incite les travailleurs déjà partiellement insérés dans l'emploi à s'y insérer davantage, mais, dans le même temps, le Gouvernement semble oublier les personnes les plus éloignées de l'emploi. Je souscris donc à l'analyse de notre collègue, pour lequel la prime d'activité, en l'espèce, est plus un soutien au pouvoir d'achat qu'une incitation à retourner vers l'emploi. S'agissant de la situation des mineurs non accompagnés, l'année dernière, un rapport d'information avec notre ancien collègue Jean-Pierre Godefroy, je demande à l'État une vraie prise en charge de cette compétence, en raison des difficultés des départements à y répondre. Depuis 2014, l'augmentation du nombre de mineurs non accompagnés est en forte hausse. Comme on l'a vu ces derniers mois, cette évolution est parfois difficile à vivre pour les départements.

je salue la proposition de Philippe Mouiller de créer un programme budgétaire distinct dédié à l'accueil des mineurs non accompagnés, obligeant l'État à assumer cette compétence. Les départements ne sont pas tous égaux pour évaluer l'âge des jeunes accueillis ou traiter les documents administratifs. C'est pourquoi je propose une plateforme à l'échelle soit régionale, soit interdépartementale, pour plus de compétence et d'équité dans l'évaluation des jeunes. Très bien ! Toutefois, l'action la plus décisive reste le renforcement de la lutte contre les filières de passeurs, en coopération avec les États d'origine des mineurs non accompagnés. Cette lutte relève de la compétence de l'État. La question reste posée : comment favoriser le développement des pays de départ pour diminuer les candidats à la migration ? J'y insiste, au-delà de la distinction entre majeurs et mineurs, le problème central demeure le même, à savoir le départ d'une population recherchant, à travers une migration, une terre d'accueil pouvant assurer la sécurité et l'autonomie financière. Enfin, je ne peux clôturer mon intervention sans évoquer la grande cause nationale du quinquennat : l'égalité entre les femmes et les hommes.

304, « Inclusion sociale et protection des personnes », se caractérise par une hausse de 14 % de ses crédits, liée à la revalorisation exceptionnelle de la prime d'activité de 20 euros pour les revenus supérieurs à 0,5 SMIC. Le Gouvernement souhaite

euros à 900 euros. Cela représente un progrès sensible. Notre groupe approuve cette mesure importante en faveur des personnes en situation de handicap.

ces mineurs, de plus en plus nombreux, sont le plus souvent dans des situations complexes et difficiles. Cette charge est de plus en plus lourde pour nos collectivités territoriales. elle sera insoutenable. L'État doit prendre sa part de responsabilités pour soutenir davantage les départements et assurer l'hébergement d'urgence et l'évaluation.

Elle se place au sixième rang des missions budgétaires de l'État. Elle est au coeur de l'action publique en matière d'attention portée aux personnes les plus en difficulté. Le groupe Les Indépendants - République et territoires se félicite de cet effort budgétaire au bénéfice des plus fragiles et

Madame la présidente, mesdames les ministres, mes chers collègues, le projet de loi de finances pour 2019 prévoit une augmentation des crédits de la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances dont le montant passera de 19,44 milliards en 2018 à 20,93 milliards en 2019, ce qui correspond à une augmentation de 7,7 %. Par les temps qui courent, c'est plutôt une bonne surprise, d'autant que la majeure partie de ces crédits est destinée à financer la prime d'activité et l'allocation aux adultes handicapés, qui relèvent toutes les deux des programmes 304 et 157. Les crédits du programme 157, « Handicap et dépendance », sont donc en hausse, ce qui s'explique essentiellement par la revalorisation exceptionnelle de l'allocation aux adultes handicapés. Si nous nous réjouissons de cette augmentation, nous déplorons la réduction du nombre de ses bénéficiaires, du fait de l'abaissement du plafond de ressources pour les couples. En outre, sa revalorisation est désindexée de l'inflation, ce qui entraînera forcément une baisse de son montant au fil du temps. En outre, cette mesure exceptionnelle ne suffit pas à faire oublier les nombreuses décisions qui ont récemment porté atteinte au pouvoir d'achat et aux conditions d'existence des personnes en situation de handicap, comme la suppression du complément de ressources ou le rejet de notre proposition de loi portant suppression de la prise en compte des revenus du conjoint dans la base de calcul de l'AAH. Concernant les crédits du programme 304, « Inclusion sociale et protection des personnes », le constat est le même : leur hausse s'explique essentiellement par la revalorisation exceptionnelle de la prime d'activité. doit être nuancée, car plusieurs mesures, telles que la baisse de l'abattement, le gel des revalorisations annuelles en fonction de l'inflation et l'exclusion des bénéficiaires de pensions d'invalidité et de rentes AT-MP restreignent la portée de cette allocation. Au fond, ce sont des augmentations de crédits en trompe-l'oeil, qui masquent, en réalité, des mesures d'économies, le Gouvernement prenant aux uns pour donner aux autres. Et votre plan Pauvreté, madame la ministre, ne nous rassure pas ! Éric Bocquet en ayant déjà parlé, je ne m'y attarderai pas. De plus, toujours dans le programme 304, les financements liés au suivi des mineurs non accompagnés progressent, mais cette augmentation des crédits est contrebalancée par le nombre croissant de bénéficiaires. La mise en oeuvre de ce dispositif dépend des départements, qui sont en grande difficulté, vu leur étranglement financier, tandis que les aides versées par l'État sont largement insuffisantes. Le Gouvernement doit prendre ses responsabilités et assurer une réelle protection de ces mineurs en danger, dont la précarité est dénoncée par de nombreuses associations.

à ces professionnels d'exercer leurs missions dans de bonnes conditions. J'en viens à présent au programme 137, « Égalité entre les femmes et les hommes ». De nouvelles actions ont été ouvertes, prévoyant notamment de favoriser l'accès aux droits pour les femmes, le développement de la culture de l'égalité et de financer les délégations régionales aux droits des femmes. Cependant, le budget correspondant, à euros constants, n'est pas suffisamment important pour mener une politique de lutte contre les inégalités ambitieuse : il ne s'élève même pas à 30 millions d'euros, soit 0,007 % du budget de la France ! Même s'il faut également prendre en compte les budgets transversaux, nous ne pouvons que constater et regretter que la prétendue grande cause du quinquennat ne bénéficie pas de moyens supplémentaires. De même, nous regrettons que, dans le nouvel intitulé des actions n 21, 22 et 23, toute référence à la lutte contre la prostitution ou à la lutte contre les violences sexistes ait totalement disparu. Nous avions été nombreuses et nombreux, lors de l'examen du PLF de l'an dernier, à intervenir sur la baisse de l'enveloppe de l'AFIS, mise en place dans le cadre des dispositifs de sortie de la prostitution. Le Gouvernement justifie la nouvelle baisse par les difficultés de mise en oeuvre sur le terrain et le peu de personnes potentiellement concernées. Nous sommes en désaccord avec ce raisonnement et pensons, au contraire, comme notre collègue Tourenne, que ce dispositif va monter en puissance, à condition que le Gouvernement le soutienne vraiment.

Alors que la France traverse une crise profonde, vous continuez d'appliquer vos vieilles recettes. Vous continuez à ne pas entendre celles et ceux qui souffrent de vos choix politiques profondément injustes et qui manifestent jour après jour. Nous voterons contre la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances » du projet

j'ai l'honneur de vous présenter, avec Sophie Cluzel, secrétaire d'État chargée des personnes handicapées, le budget de la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances souligner d'emblée la cohérence politique de ce budget avec le projet de loi de financement de la sécurité sociale : ils portent les mêmes choix et les mêmes priorités. D'abord, priorité est donnée aux personnes les plus fragiles, afin de répondre de façon spécifique à leurs attentes prioritaires et d'agir sur les facteurs du déterminisme social. est également donnée aux salariés les plus modestes, pour que le travail paie davantage. Cette priorité sociale du Gouvernement se lit d'abord dans l'évolution des crédits de la mission, qui augmentent de 7 %.

Ce budget est d'abord celui d'une solidarité renforcée, au bénéfice de nos concitoyens les plus fragiles. Je veux évoquer, en premier lieu, la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté, que nous avons présentée le 13 septembre dernier. il s'agit d'une politique ambitieuse et globale, qui vise à éviter que les enfants pauvres d'aujourd'hui ne deviennent les adultes pauvres de demain. Le Gouvernement a bâti une stratégie qui va se déployer dans tous les territoires et qui a pour objectifs de renforcer l'accès aux services de la petite enfance, de conforter les droits fondamentaux des enfants et de renforcer l'insertion des jeunes Le programme 304 est le support budgétaire principal de cette stratégie. Il porte les crédits dédiés à la contractualisation avec les territoires à hauteur de 171 millions d'euros en 2019. 135 millions d'euros seront consacrés à la contractualisation avec les départements, laquelle portera sur les quatre objectifs suivants : l'accompagnement des sortants de l'aide sociale à l'enfance, le renforcement de l'accompagnement des bénéficiaires du RSA, la formation des travailleurs sociaux et l'accueil social de proximité. L'effort de solidarité s'exprime également et fortement au travers de l'évolution des crédits du programme 157, Handicap et dépendance », qui sont portés à 11,9 milliards d'euros, soit une augmentation de 5,1 %. Cette hausse très importante traduit la priorité, pour le quinquennat, que constitue la construction d'une société plus inclusive. Elle permet de concrétiser l'engagement du Président de la République en faveur de la revalorisation de l'allocation aux adultes handicapés, afin de donner à tous leur juste place dans le projet national et de garantir un revenu minimal aux personnes dont le handicap interdit ou limite fortement l'accès au travail. La revalorisation de l'AAH a porté, le mois dernier, le niveau de l'aide à taux plein à 860 euros, ce qui représente une progression de 41 euros par mois.

Parce que le travail conduit à l'émancipation sociale, le soutien à l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés est également renforcé, notamment dans le milieu ordinaire, avec un effort important en faveur de l'emploi accompagné. Ce dispositif combine accompagnement médico-social et accompagnement professionnel pour les travailleurs handicapés. Les crédits dédiés à ces emplois accompagnés augmenteront ainsi de 40 % par rapport à l'année précédente. L'engagement du Gouvernement s'inscrit pleinement dans le cadre du comité interministériel du handicap organisé le 25 octobre dernier, qui a permis de mobiliser l'ensemble des ministères autour du Premier ministre, Édouard Philippe, et de la secrétaire d'État, Sophie Cluzel, pour mettre en oeuvre des mesures de simplification en faveur des en faveur des droits des personnes et lutter contre les ruptures de parcours des personnes handicapées. L'effort de solidarité bénéficie, en troisième lieu, à nos compatriotes d'outre-mer, dans deux territoires confrontés à des difficultés sociales très importantes : la Guyane et Mayotte. Conformément à l'engagement pris par le Président de la République en octobre 2017, l'État reprend à sa charge le financement du RSA dans les deux collectivités de Guyane et de Mayotte à compter du 1 janvier 2019, pour un montant de 170 millions d'euros. Il s'agit de soulager ces collectivités du poids du financement et de l'attribution du RSA, sans pour autant remettre en cause leurs compétences pour ce qui concerne l'insertion des bénéficiaires. l'État assume pleinement ses responsabilités au sujet des mineurs non accompagnés. Le Gouvernement a bien entendu les difficultés des départements, et il a fait le choix de renforcer le soutien qu'il leur apporte, à deux niveaux complémentaires : d'une part, pour la mise à l'abri et l'évaluation des personnes se présentant comme mineures- à compter de 2019, l'appui financier de l'État sera renforcé par une compensation plus juste des dépenses engagées, sur la base d'un forfait par jeune réévalué d'autre part, l'État prendra en charge une partie des dépenses supplémentaires des départements au titre de l'aide sociale à l'enfance, l'ASE, lorsque les personnes sont effectivement évaluées comme mineures. Pour la seconde année consécutive, un dispositif exceptionnel sera mis en oeuvre en 2019. Je tiens à insister particulièrement sur ce second volet. à l'issue d'échanges très nourris et étroits avec l'Assemblée des départements de France, l'ADF, le Gouvernement a souhaité aller plus loin que ce qui était prévu. Il a ainsi décidé de relever son concours financier. Concrètement, en 2019, une aide forfaitaire de 6 000 euros sera octroyée aux départements pour 75 % des mineurs non accompagnés supplémentaires admis à l'ASE par rapport à l'année précédente, contre 50 % auparavant. En tout, ce sont plus de 175 millions d'euros qui seront consacrés, en 2019, au soutien des départements. Plus largement, l'effort engagé à la fois dans le cadre de la stratégie Pauvreté et pour la gestion des mineurs non accompagnés traduit la volonté du Gouvernement d'oeuvrer à l'avènement d'une nouvelle contractualisation entre l'État et les conseils départementaux dans la déclinaison des politiques sociales. Je mènerai cette politique de concert avec Jacqueline Gourault, ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. La mission « Solidarités » porte également un effort sans précédent au bénéfice des salariés modestes de ce pays. La prime d'activité bénéficie aujourd'hui à 2,8 millions de nos concitoyens. C'est une prestation importante : elle soutient le pouvoir d'achat et incite à la reprise d'activité. République a pris l'engagement de la revaloriser de 80 euros pour un salarié au SMIC d'ici à la fin du quinquennat. Cette revalorisation s'ajoutera au gain de pouvoir d'achat de 20 euros par mois du fait de la suppression des cotisations salariales maladie et chômage, laquelle est pleinement effective depuis le mois d'octobre

plus important et plus rapide que prévu par la loi de programmation des finances publiques. En outre, cette prime augmentera de nouveau de 20 euros en 2020 et de 20 euros en 2021, soit un total de 80 euros d'ici à 2021. les sénateurs, le montant des crédits consacrés à la prime d'activité était seulement de 4,3 milliards d'euros en loi de finances initiale pour 2017 deux ans après, parce que nous avons rétabli la sincérité budgétaire, parce que le montant de la prime d'activité progresse et parce que le nombre de bénéficiaires augmente, ce montant dépasse 6 milliards d'euros. Cet effort exceptionnel est le signe tangible de la priorité qu'accorde le Gouvernement au pouvoir au pouvoir d'achat des travailleurs aux revenus modestes. J'évoquerai à présent un programme à forte dimension transversale, le programme 137. Comme vous le savez, l'égalité entre les femmes et les hommes a été érigée par le Président de la République en grande cause nationale du quinquennat.

Le programme 137 est l'un des outils de cette politique, qui mobilise un ensemble de crédits beaucoup plus important. Si le montant de ce programme n'augmente pas, le taux d'exécution des crédits est en hausse de plus de trente points.

des tribunaux du contentieux de l'incapacité, les TCI, et d'une partie des commissions départementales d'aide sociale, les CDAS, vers les futurs pôles sociaux des tribunaux de grande instance. Cette réforme prendra effet le 1 janvier 2019. Son application sera assurée grâce à la mise à disposition du ministère de la justice des personnels qui travaillent dans ces tribunaux et qui relèvent soit des organismes de sécurité sociale, soit du ministère des solidarités et de la santé, ainsi que des moyens de fonctionnement associés.

au sein du ministère de la justice. En conséquence, nous proposons un transfert supplémentaire d'emplois du programme 124 vers le programme 166, à hauteur de 5 ETPT, représentant un coût chargé de 341 362 euros.

Nous vous encourageons donc à veiller à préserver le montant de crédits satisfaisant pour le bon fonctionnement des ministères sociaux ; étant donné que vous en êtes les garantes, nous émettons un avis favorable sur cet amendement.

Il s'agit de consacrer par la loi ce qui n'existe pour l'heure qu'au sein des programmes annuels de performance et n'a donc pas de valeur contraignante. Il s'agit surtout d'envoyer un signal fort à l'État au sujet de cette mission : les conseils départementaux ont toujours estimé qu'elle relevait de sa compétence exclusive, au titre de la politique migratoire,

La maquette actuelle du programme 304, « Inclusion sociale et protection des personnes », est issue de la fusion, en 2015, de l'ancien programme 304, « Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales et du programme 106, « Actions en faveur des familles vulnérables », dont relevait alors le dispositif d'évaluation et de mise à l'abri des mineurs non accompagnés. Cette évolution de périmètre a permis d'établir un cadre budgétaire plus lisible pour les politiques publiques de la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances De plus, elle s'inscrit pleinement dans la ligne tracée par le comité interministériel pour la modernisation de l'action publique, lequel plaide pour une réduction du nombre de programmes.

d'assumer les conséquences des politiques qu'il conduit ou ne conduit pas. Or les dépenses en question sont considérables. Mme la ministre nous assure que l'effort a augmenté : certes

Madame la ministre, vous vous dites troublée par les propos de mon collègue Jean-Louis

Tourenne. Madame la ministre, nous regrettons profondément que les ministères sociaux fassent partie des ministères non prioritaires dans la politique actuellement menée. Touchés de manière importante par les mesures d'économies budgétaires, ces ministères pâtissent des décisions prises par votre gouvernement.

des mineurs non accompagnés. Dans le département que j'ai présidé, ils avaient le même statut que tous les autres enfants, ils coûtaient le même prix et ils étaient pris en charge dans les meilleures conditions humaines, qui leur permettaient, d'ailleurs, d'obtenir ensuite des contrats jeune majeur ! S'il vous plaît, ne venez pas me donner de leçons à cet

générale de l'État, qui a été annoncée et qui est nécessaire pour réduire la dépense publique. Néanmoins, nous sommes très attentifs à ce qu'elles

femmes ». La refonte de la présentation budgétaire que vous nous proposez cette année sert en effet à masquer une diminution des crédits de 1 million d'euros à périmètre constant, dont 900 000 euros sur l'accompagnement des personnes prostituées qui s'engagent dans le parcours de sortie de la prostitution. C'est pourquoi nous souhaitons, par cet amendement, rétablir les crédits de cette mission essentielle qu'est l'accompagnement et la protection des victimes du proxénétisme au niveau qui était le leur avant que cette majorité parlementaire ne s'installe.

cette baisse concerne surtout l'aide financière à l'insertion sociale et professionnelle, l'AFIS, les crédits nationaux et déconcentrés dévolus aux associations étant relativement préservés.

nous apportons un soutien de 2,1 millions d'euros aux associations chargées d'accompagner les personnes en situation de prostitution. Par ailleurs, 2 millions d'euros de crédits sont destinés à l'aide financière d'insertion sociale et professionnelle, dont on sait que la montée en charge a été assez lente.

Au 31 août 2018, il y avait 68 bénéficiaires et 85 personnes engagées dans un parcours de sortie de prostitution ; 35 commissions chargées de délivrer l'AFIS

de façon sincère la montée en charge progressive d'un dispositif dont on connaît la complexité, car il s'adresse à des personnes très éloignées et en situation très précaire. Nous travaillons pour accompagner au mieux les associations, qui font un travail absolument remarquable sur le terrain. Je le répète, c'est un budget sincère.

je suis toujours très circonspect devant les discours qui revendiquent la sincérité de manière tellement réitérée.

sans restreindre les actions que vous allez mener. S'agissant de cet amendement, il a le même objet que le précédent : le droit des personnes prostituées à sortir du système prostitutionnel semble gravement menacé par la restriction des crédits. Un signal politique fort en faveur de l'abolition est indispensable, pour continuer à affirmer que le corps des femmes n'est pas à vendre. Le projet de loi de finances pour 2019 en offre l'occasion et nous devons la saisir. Le présent amendement vise ainsi à réinjecter les 900 000 euros manquants à la mise en oeuvre de l'accompagnement des personnes prostituées vers l'insertion sociale et

parole est à M. Jean-Louis Tourenne. C'est un ! Nous nous inquiétons de l'absence de budget affecté pour 2019 aux têtes de réseaux, qui font un travail remarquable au quotidien sur nos territoires pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles et pour accompagner les personnes qui en sont victimes. Alors que 500 000 euros leur étaient consacrés depuis plusieurs années dans le projet de loi de finances, aucune affectation budgétaire précise n'est donnée pour 2019. Cela provoque, dans les réseaux, une vive inquiétude, que nous partageons, car, sans ces budgets, plusieurs d'entre eux ne seront plus en capacité d'exercer leur mission d'intérêt général et devront tout simplement mettre la clé sous la porte.

indispensable. C'est pour moi un moyen d'attirer l'attention sur des nécessités et sur le fait que les baisses constatées seront largement préjudiciables aux politiques qui devraient être menées en faveur de la lutte contre la prostitution.

En France, les protections hygiéniques représentent un budget annuel allant, selon les sources, de 25 euros à plus de 50 euros par femme. Une femme utilise en moyenne 22 tampons ou serviettes par cycle, ce qui représente un coût estimé entre 1 500 euros au cours de sa vie. Certaines mutuelles, notamment étudiantes, se sont d'ores et déjà emparées de ce problème sanitaire et social, et proposent un forfait de 20 euros à 25 euros par an pour le remboursement de ces protections, sur présentation du ticket de caisse ou d'une facture.

à satisfaire ce besoin de protection des plus élémentaires. À la rue ou en centre d'hébergement, les règles restent souvent un moment pénible, humiliant et très difficile à gérer pour beaucoup contraintes parfois à utiliser des morceaux de vêtements pour se protéger. Le sujet touche aussi nos adolescentes : certaines jeunes filles manquent l'école, car elles n'ont pas accès aux protections hygiéniques qui leur permettraient de s'y rendre pendant leurs règles. À ce sujet, je tiens à saluer l'action de l'association Règles élémentaires, fondée en 2015 par Tara Heuzé, qui organise des collectes de serviettes hygiéniques. Grâce à cette association, Grâce à cette association, plus de 200 000 protections hygiéniques ont été distribuées gratuitement en France depuis trois ans. Face à ces enjeux sanitaires et de dignité, le présent amendement vise à expérimenter, au sein de régions volontaires, idéalement en métropole et outre-mer, la libre distribution de protections hygiéniques dans différents lieux accueillant, notamment, des publics vulnérables.

pour les personnes les plus sévèrement handicapées, adopté en 2005. Le Gouvernement entend ainsi rationaliser les prestations complémentaires de car la coexistence du complément de ressources- 179,31 euros par mois -et de la majoration pour la vie autonome- 104,77 euros par mois -nuirait à la lisibilité de l'AAH. Il estime donc que la fusion de ces deux compléments de ressources répond à une nécessaire simplification du dispositif et qu'elle permettra d'alléger les démarches des bénéficiaires de l'AAH. de l'AAH. Elle lui permettra également, toutefois, de les aligner sur la prestation la moins coûteuse, la majoration pour la vie autonome, par ailleurs elle-même soumise à la condition de percevoir une aide au logement. Le Gouvernement fera ainsi des économies de l'ordre de 75 euros à 179 euros par mois par personne concernée. en décembre 2016, on comptait 152 883 bénéficiaires de la majoration pour la vie autonome et 68 118 bénéficiaires bénéficiaires du complément de ressources. Le Conseil national consultatif des personnes handicapées, le CNCPH, a exprimé son vif refus de cette mesure, rappelant que les deux compléments à l'AAH, s'ils ont effectivement des caractéristiques communes, ont également des motifs distincts : le complément de ressources a pour objectif de compenser l'absence durable de revenus d'activité des personnes qui sont dans l'incapacité de travailler, alors que la majoration pour la vie autonome favorise l'accès des personnes en situation de handicap à un logement autonome, sur la base d'un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 %.

La pauvreté des personnes en situation de handicap, des bénéficiaires de l'AAH, d'une pension d'invalidité ou d'une rente, ou encore des travailleurs handicapés est une réalité prégnante sur laquelle je refuse de fermer les yeux. C'est pourquoi je soutiendrai la demande de suppression de cet article.

Nous considérons que ces arguments ne sont pas recevables, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, ce complément de ressources constituait une avancée permise par la loi du 11 février 2005, laquelle avait mis en place une garantie de ressources pour les personnes les plus sévèrement handicapées. Ensuite, bien que ces deux compléments de l'AAH partagent des similarités, ils ont des caractéristiques propres : le complément de ressources a pour objectif de compenser l'absence durable de revenus d'activité des personnes qui sont dans l'incapacité de travailler

qui gèrent plus de 4 millions de demandes par an et traitent automatiquement et simultanément les demandes de complément de ressources et d'allocation aux adultes handicapés.

La suppression du complément de ressources au profit de la majoration pour la vie autonome est une mesure de simplification importante, qui évitera de soumettre le demandeur à une double appréciation de son taux d'incapacité permanente, d'une part, et de sa capacité minimale de travail, d'autre part. C'est pour arrêter de demander aux personnes d'apporter constamment la preuve de leur handicap que le Premier ministre a décidé, notamment, de rendre possible l'attribution des droits à vie, dans le cadre du dernier comité interministériel du handicap, le 25 octobre dernier. À vrai dire, le maintien du complément de ressources est une survivance historique : il aurait dû disparaître avec la création, en 2005, de la prestation de compensation du handicap, la PCH. la PCH. Destinée à soutenir l'autonomie des personnes handicapées à domicile, cette prestation bénéficie aujourd'hui à plus de 280 000 personnes, pour un montant de près de 2 milliards d'euros. janvier 2020, du complément de ressources au profit de la majoration pour la vie autonome est organisée de manière à préserver strictement les droits des bénéficiaires actuels. Ils continueront d'en bénéficier, y compris lorsqu'ils formuleront une demande de renouvellement, pendant une durée de dix ans. Au-delà de cette mesure, je veux rappeler que le Gouvernement soutient résolument l'autonomie dans le logement des personnes en situation de handicap, au travers notamment de l'habitat inclusif, auquel la loi ÉLAN, récemment adoptée, donne une définition législative.

de remise à plat de la prestation de compensation du handicap, dans le cadre de la conférence nationale du handicap 2018-2019 lancée lundi dernier, 3 décembre, journée internationale des personnes handicapées. Respectueuse de la responsabilité particulière des départements dans ce domaine, j'ai confié le pilotage de ce chantier à Mme Marie-Pierre Martin, première vice-présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire. Vous pouvez compter sur ma détermination pour aboutir à de véritables

Nous l'avons combattue, mais nous n'avons pas été entendus. Nous le savons : s'il n'y a pas d'obligation dès le départ, les choses ne se feront pas. En effet, aménager des logements existants pour des personnes handicapées,

En application de l'article 4 de la loi n° 2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, l'article 621-1 du code pénal dispose que l'outrage sexiste est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe et précise les circonstances aggravantes pour lesquelles il est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Ce dispositif a vocation à réprimer le harcèlement dans l'espace public, c'est-à-dire un comportement qui contrevient à l'égalité entre les femmes et les hommes et à la liberté de circulation des femmes. Il s'agit,, de changer ce type de comportement.

ainsi que la lutte contre les violences sexuelles et sexistes.

Le législateur a prévu qu'un rapport sur la politique publique de lutte contre les violences sexuelles et sexistes dont sont victimes les enfants, les femmes et les hommes serait élaboré. Ce rapport devra notamment récapituler, par ministère et pour le dernier exercice connu, l'ensemble des crédits affectés à cette politique publique, évaluer au regard des crédits affectés la pertinence des dispositifs de prévention et de répression de ces violences. Il comportera une présentation stratégique assortie d'objectifs et d'indicateurs de performance, une présentation des actions ainsi que des dépenses et des emplois avec une justification au premier euro. Tous les éléments

de personnel déstabilisée du fait du choix laissé aux agents de l'État de ne pas rejoindre leur nouvelle affectation en MDPH, mais de regagner leur administration d'origine. L'État n'ayant pas toujours été en mesure de remplacer physiquement les intéressés, les MDPH ont dû pourvoir aux vacances par le recrutement d'agents contractuels.

ou remplaçants nécessaires. Ainsi, de 2014 à 2016, les dépenses de personnel réglées directement par les MDPH ont crû de 12,4 %. Or, contrairement aux collectivités territoriales et à leurs régies, les GIP MDPH employeurs ne sont pas exonérés de taxe sur les salaires ; ils sont soumis, dans ce domaine, au même régime que les entreprises privées. Le présent amendement vise à les exonérer de cette taxe, afin de préserver leur situation financière fragile.

Toutefois, instaurer une exonération pour les groupements d'intérêt public MDPH ne nous paraît pas justifié, car ces établissements dotés de la personnalité morale relèvent de la catégorie des établissements redevables de la taxe sur les salaires, comme les établissements publics ou les organismes médico-sociaux.

car accorder une exonération de taxe sur les salaires aux seuls GIP MDPH employeurs serait contraire au principe d'égalité devant la loi et susciterait des demandes tout aussi légitimes de la part d'autres structures du secteur médico-social.

Ainsi, comme tous les groupements d'employeurs, les GIP MDPH sont redevables de la taxe sur les salaires pour leurs personnels contractuels si moins de 90 % de leurs recettes ont été soumises à la TVA au titre de l'année précédente. En revanche, la taxe sur les salaires ne s'applique pas aux rémunérations des personnels de l'État ou des collectivités territoriales mis à leur disposition et qui restent rémunérés par leur administration ou leur collectivité. Réserver une exonération de taxe sur les salaires aux GIP MDPH poserait une difficulté sur le plan du principe d'égalité devant la loi. En effet, ces structures ne sont pas les seules du secteur médico-social et ne sont pas placées dans une situation différente des autres personnes morales chargées de la gestion d'un service public dans le domaine social. Cette mesure, si elle était adoptée, susciterait donc des demandes également justifiées de la part des autres acteurs du secteur médico-social, auxquelles il serait très difficile de ne pas donner une suite favorable.

Cette simplification et les droits à vie allégeront la charge des personnels. Par ailleurs, je tiens à vous signaler que, parmi les cinq chantiers que nous avons ouverts lors de la conférence nationale du handicap,

belles déclarations, les bonnes intentions, on n'arrive pas à changer les choses, parce qu'on a créé une sorte de droit acquis et que ceux à qui on voudrait retirer cet avantage manient immédiatement la menace.

en appui de cette transformation. Vous pouvez compter sur ma détermination, et je veux bien compter sur votre appui : réfléchissons ensemble à l'amélioration et à la rénovation de ces dispositifs indispensables

Nous envisageons une expérimentation de la carte dématérialisée, qui ne pourra pas se faire partout sur le territoire, notamment en Guyane. Cette expérimentation est en train d'être organisée.

jusqu'au 31 décembre 2024 pour les seules personnes ayant bénéficié au moins une fois du dispositif entre le 31 décembre 2017 et le 31 décembre 2018. Nous ne pouvons qu'être favorables à cet article, qui sécurise la situation des bénéficiaires de 2018 à 2024.

D'abord, vous mettez en oeuvre un droit à deux vitesses : des personnes placées dans des situations équivalentes auront des droits différents. Ensuite, vous sanctionnez le non-recours, en contradiction avec l'objectif que vous avez annoncé de lutter contre le non-recours aux droits. Les personnes qui n'ont pas demandé la prestation entre fin 2017 et fin 2018, alors qu'aucune campagne d'information particulière n'a été menée par le Gouvernement, en seront définitivement privées dans les années à venir.

qu'il invoque notamment- à tort -pour légitimer la suppression du complément de ressources. Cette situation est d'autant plus regrettable que les bénéficiaires du dispositif forment un public particulièrement vulnérable.

spécial. Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le président de la commission des affaires sociales, mes chers collègues, le projet de loi de finances prévoit cette année une augmentation de 3,5 % des crédits de la mission « Santé », après une hausse inédite de 10 % en loi de finances pour 2018. Le budget de la mission atteindra donc 1,423 milliard d'euros en 2019.

Cette année encore, madame la ministre, vous diminuez le budget alloué aux opérateurs sanitaires pour compenser l'augmentation des crédits dédiés au programme 183, c'est-à-dire essentiellement à l'aide médicale de l'État. Au total, les crédits du programme 204 ont diminué de 25 % depuis 2013, alors que ceux du programme 183 ont progressé de 27 % sur la même période.

parlons, une réforme de l'AME est absolument incontournable. C'est ce que pense la commission des finances du Sénat, qui préconise un resserrement du dispositif d'accès aux soins

J'espère que vous nous entendrez cette année, madame la ministre. Par ces deux amendements, la commission des finances affirme sa volonté de réformer en profondeur l'AME, afin de ramener cette dépense à un niveau plus soutenable.

la prévention s'impose désormais comme le maître mot des annonces gouvernementales dans le domaine de la santé. Mais, pour ce qui est des moyens, les intentions peinent encore à se matérialiser. En effet, si les crédits de la mission « Santé » progressent globalement de 3,4 %, c'est exclusivement le fait de l'augmentation des moyens de l'AME. Les crédits du programme 204, « Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins », diminuent de 1 %. En leur sein, les moyens des agences sanitaires sont au mieux stabilisés. Le renforcement du pilotage de l'État au travers de la mise en place du Comité d'animation du système d'agences constitue un progrès, mais les marges de manoeuvre de l'Agence nationale de sécurité En particulier, à la suite de la polémique autour du fonctionnement du registre des malformations congénitales « REMERA » en Rhône-Alpes, la commission des affaires sociales souhaite attirer votre attention, madame la ministre, sur les besoins de professionnalisation de nos réseaux décentralisés de surveillance sanitaire. Il est nécessaire de renforcer leur coordination et leur évaluation scientifique sous l'égide de Santé publique France et de l'ANSES. La commission des affaires sociales s'est également émue de la fragilité du financement du volet « recherche » des plans de santé médicale, participe ainsi à de nombreux plans de santé publique, dont les plans Autisme et « Maladie de Lyme », pour lesquels les cohortes sont prêtes. Seul problème, les opérations ont dû être retardées dans l'attente des fonds nécessaires. 17 millions d'euros a finalement été annoncée pour la recherche en santé publique : madame la ministre, pouvez-vous nous confirmer que ces crédits seront pérennisés dans le cadre d'un programme national de recherche en santé publique, présenté en loi de finances ? Je sais que ce sujet ne relève pas directement de votre ministère, mais vous pouvez au moins solliciter Quelle part le ministère de la santé prendra-t-il dans le pilotage de ces crédits ? Enfin, la commission a rappelé son attachement au maintien des crédits de l'AME. Ce dispositif humanitaire répond à une vraie exigence de santé publique, en prenant en charge des personnes démunies dont l'état de santé est souvent fortement dégradé. Nous ne pouvons donc pas souscrire à la proposition de la commission des finances de minorer les crédits du programme 183, « Protection maladie », ou de réintroduire un droit de timbre. Nous ne ferions qu'aggraver leur état de santé et prendrions le risque d'engorger à terme les services d'urgence hospitaliers. Sous réserve de ces observations, la commission a émis un avis favorable à l'adoption des crédits de la mission « Santé » du projet de loi de finances pour 2019. Mes chers

développer la politique de prévention, assurer la sécurité sanitaire, organiser une offre de soins de qualité adaptée et volontaire, qui tienne compte des spécificités de chaque territoire. Pour préserver un système de santé dont nous pouvons et devons être fiers, le Gouvernement est déterminé, dans le cadre de la stratégie nationale de santé et du plan « Ma santé 2022 », à mobiliser tous les acteurs pour réduire les inégalités qui demeurent, consolider le système de prise en charge solidaire par une vision coordonnée du système de santé, et ce dans le cadre d'une logique de parcours intégrant la promotion de la santé et la prévention. Vous le savez, les crédits de la mission « Santé » ne constituent qu'une partie des moyens de notre politique publique sanitaire. Pour mémoire, l'objectif de dépenses de la branche maladie, maternité, invalidité et décès

Pour 2019, le projet de loi de finances fixe les crédits de la mission « Santé » à 1,422 milliard d'euros, en hausse de 3,4 %. L'importance de cette mission, tant dans sa structure que dans les objectifs qu'elle fixe, implique qu'on la regarde dans le détail. Elle comporte deux programmes, le programme 204 et le programme 183. Les crédits du programme 204 relatifs à la prévention, la sécurité sanitaire et l'offre de soins sont quasi stables après avoir enregistré une hausse de 10 % en 2018. Ce programme, qui représente 34 % des crédits de la mission, retrace en particulier les subventions pour charges de service public versées à des opérateurs sanitaires de l'État. En 2019, la réflexion sera poursuivie en liaison avec chacun des opérateurs, afin d'améliorer leur pilotage, de favoriser leur pleine contribution aux efforts requis dans le cadre de la programmation pluriannuelle des finances publiques pour la période 2018-2022, le tout dans une volonté de mieux mutualiser et rationaliser, afin de mieux servir tout en dépensant moins. Les crédits du programme 183 relatifs à la protection maladie des publics les plus défavorisés et des victimes de l'amiante progressent,

Dans ce programme, les dépenses prévisionnelles pour l'AME sont en augmentation de 45 millions d'euros. Elles s'élèvent à 935 millions d'euros, afin de répondre non seulement au problème récurrent de sous-budgétisation, mais également à un objectif humanitaire et sanitaire. Je le rappelle, le principe de l'AME est essentiel. Premièrement, il répond au besoin de soigner les gens en première nécessité. Le serment d'Hippocrate n'est pas négociable : pour le médecin, soigner sera toujours un devoir. Deuxièmement, il répond à une préoccupation de santé publique, en particulier, la lutte contre les maladies infectieuses et les maladies de la précarité, la tuberculose, la gale et bien d'autres maladies, qui peuvent toucher non seulement l'individu, mais aussi son entourage et, en conséquence, une partie de la population. Mes chers collègues, certains d'entre vous ont la conviction que l'AME est un coût pour l'État et, donc, pour nos concitoyens. Seulement, les maladies contagieuses ne choisissent ni leur pays ni l'origine de celui qui sera contaminé. Alors, à défaut de voir cette volonté comme une démarche humanitaire, faites-le pour vous et pour votre entourage, afin de vous protéger en évitant une contamination par autrui. Le virus ne s'interroge pas sur la nationalité : toute personne pour lui est un vecteur de transmission de la maladie, ni plus ni moins. Décider de protéger ces femmes et ces hommes n'empêche en rien une politique de contrôle et de lutte contre la fraude. Elle sera renforcée, afin que la mise en oeuvre de la solidarité nationale s'accompagne d'une gestion rigoureuse du dispositif. Pour ce faire, l'instruction des demandes d'AME sera centralisée en 2019 autour de trois caisses pivot, à Paris, Bobigny et Marseille, et des procédures harmonisées seront mises en place. Sans AME, notre territoire prendrait le risque de la contagion et d'une renaissance de certaines maladies. L'AME est un acte humanitaire de base, au même titre qu'un acte de prévention nationale. Avant de conclure, permettez-moi de revenir sur les litiges amiables et contentieux mis à la charge de l'État au titre d'accidents médicaux. Si, depuis deux ans, le nombre de demandes d'indemnisation des victimes de l'amiante tend à diminuer, d'autres drames de santé publique méritent toute notre attention. En 2016, les parlementaires ont posé les bases du dispositif d'indemnisation des victimes du valproate de sodium ou de ses dérivés. Les instructions des demandes d'indemnisation des victimes sont confiées à l'Office national d'indemnisation Pourtant, un problème persiste : le processus d'indemnisation se met en place plus rapidement que les nouvelles découvertes sur les mécanismes d'intoxication médicamenteuse n'émergent. Par conséquent, certaines victimes déboutées dans un premier temps pourraient voir aboutir leur demande aujourd'hui.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, la mission « Santé », d'un budget de 1,8 milliard d'euros, complète les politiques de la sécurité sociale en faveur de l'accès aux soins des publics les plus défavorisés

qui prévoit une diminution de 3,8 milliards d'euros des dépenses de santé et la non-compensation des exonérations de cotisations sociales par l'État à hauteur de 2,1 milliards d'euros,

plus supportées- à juste titre -par nos concitoyennes et nos concitoyens, et qu'entre 5 et 9 millions de personnes vivent actuellement sous le seuil de pauvreté, vous diminuez les crédits destinés à la santé des populations en difficulté. C'est un non-sens Vous ne pouvez pas continuer à augmenter les cadeaux pour les plus riches et, dans le même temps, diminuer les crédits destinés aux plus précaires. De la même manière, le programme 204 considère le réseau associatif comme « un partenaire essentiel à la réalisation des priorités de santé publique », pour reprendre vous avez décidé de supprimer les contrats aidés financés pour partie par l'État, qui étaient indispensables au bon fonctionnement de la majorité des associations. Vous n'êtes pas, hélas, à une contradiction près. Ainsi, alors que la COP24 rappelle aux États les engagements pris lors de la Conférence de Paris

C'est une hérésie ! La santé environnementale doit être une priorité pour les pouvoirs publics et votre gouvernement devrait en tirer les conséquences en dégageant des moyens à la hauteur des enjeux. Pour l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, l'ANSM, dont les missions ne font que s'élargir et qui a connu une diminution de 20 millions d'euros de son budget depuis 2012, soit 13 %, de ses crédits, vous prévoyez la suppression de 23 postes pour 2019 et autant en 2020.

aux crises de la Dépakine, du Levothyrox, de l'Agréal, du laboratoire Biotrial, de l'Androcur, et compte tenu de la pénurie de médicaments ? Par ailleurs, alors que la prévention des maladies chroniques, qui touchent 15 millions de personnes en France, est une priorité du plan « Ma santé 2022 », les crédits diminuent eux

de la Dépakine ? Surtout, que prévoit le Gouvernement pour faire face aux demandes qui risquent d'être déposées par toutes les victimes potentielles de la Dépakine, dont le nombre est estimé entre 16 000 et 30 000 ? À cette baisse injustifiable s'ajoute la complexité du système pour les victimes qui doivent constituer des dossiers extrêmement lourds de déposer une demande d'indemnisation. Il faut revoir l'ensemble du système et nous donner les moyens financiers d'y parvenir. Nous aurons l'occasion d'y revenir lors de l'examen de l'article 81 et de l'amendement du Gouvernement tendant à insérer un article additionnel après ce même article.

doivent être intégrées au régime général de la sécurité sociale. Cela s'inscrit dans le prolongement de notre combat humaniste, solidaire et universel, qui refuse d'opérer des distinctions selon les nationalités, d'autant que les bénéficiaires actuels de l'AME sont pour 21 % d'entre eux des mineurs,

l'illustrent parfaitement. Le fait que le reste des crédits non réservés aux agences, qui voient leurs moyens au mieux stabilisés, soit en fait principalement consacré aux frais de justice, notamment pour l'indemnisation des accidents médicamenteux, affaiblissement du pilotage politique par le ministère ou de l'étatisation de l'assurance maladie, dont le paritarisme relève d'ailleurs davantage d'une fiction que de la réalité ? En tous les cas, il devient de plus en plus difficile de déceler une vision stratégique dans le périmètre du programme 204.

de finances pour 2019 confirme l'absence de traduction des ambitions affichées dans le plan « Priorité prévention ». En matière de prévention des addictions, c'est même un jeu à somme négative. Vous avez baissé de 13 % ces crédits, ainsi que de 28 % les crédits dévolus aux partenariats associatifs, alors que nous savons tous que, dans ce domaine, le tissu des acteurs associatifs est dense, expérimenté et précieux. rattacher ces baisses de crédits à la transformation de l'ancien fonds de prévention contre le tabac en un fonds dédié à l'ensemble des addictions à des substances psychoactives. de loi de financement de la sécurité sociale, cette extension du périmètre d'action du fonds ne s'accompagne malheureusement pas d'une augmentation de son enveloppe budgétaire, difficilement maintenue autour de 100 millions d'euros. C'est trop peu, beaucoup trop peu, alors que nous savons que le coût social et sanitaire du seul alcool s'élève à 120 milliards d'euros. Je dirai également quelques mots sur l'épidémie de VIH, dont le niveau actuel, qui s'établit à 6 000 nouvelles contaminations par an, nous engage collectivement. Nous accueillons favorablement l'augmentation de près de 6 % des crédits consacrés à cette cause. Les efforts doivent se concentrer sur l'intensification du dépistage dans les populations clés. Nous nourrissons à ce sujet une ambition réaliste si la volonté politique et les moyens suivent, celle de vaincre, pour la première fois dans l'histoire de la médecine, un virus sans vaccin. Nous savons que vos engagements en la matière sont réels et nous les saluons. La bataille en matière de prévention se mène aussi sur le front de l'environnement. Mais, avec des crédits en baisse de 20 %, les promesses de faire de la santé environnementale une priorité laissent un goût de déception. Cette diminution nous inquiète à l'approche de la révision, l'an prochain, du quatrième plan national santé-environnement et de la présentation de la nouvelle stratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens. Vous le savez, les progrès de la santé humaine dans les décennies à venir viendront, pour une part importante, de notre capacité à réduire efficacement les facteurs environnementaux qui dégradent Les enjeux sont considérables, et l'attention de nos concitoyens va croissant. La crédibilité de nos institutions sanitaires a été mise à mal à la suite de l'affaire médiatisée des malformations congénitales dans l'Ain, en Bretagne et dans les Pays de la Loire.

Cela passe par un renforcement budgétaire, notamment pour garantir la pérennité de registres de données environnementales et sanitaires, mais également par une réévaluation des méthodes d'expertise héritées de l'infectiologie et, parfois, peu adaptées aux enjeux environnementaux. De manière plus générale, l'État doit prendre ses responsabilités sur le pilotage opérationnel d'une politique de santé environnementale à part entière, impulsée à la bonne échelle, au travers des services déconcentrés de l'État, et déployée de concert avec les collectivités territoriales. Une politique de santé environnementale, oui ! Avec les collectivités territoriales, oui ! Sans le ministère, non ! J'en viens au programme 183 et à l'aide médicale de Le budget qui nous est présenté est sincère et reflète les efforts entrepris pour rendre la gestion de l'AME plus efficiente. L'alignement de la tarification des séjours hospitaliers pour les soins somatiques des patients accueillis au titre de l'AME a notamment permis des économies estimées entre 80 millions et 140 millions d'euros par an, et les efforts de rationalisation dans la gouvernance ont renforcé, à la fois, le pilotage du dispositif et le contrôle des dossiers. Ces réformes, conformes à ce que préconisait l'Inspection générale des finances dans son rapport de 2010, montrent qu'une mutualisation avec les services de l'assurance maladie engendre des économies d'échelle et va donc dans le sens d'une plus grande efficience.

encore tentés de voir le dispositif supprimé ou réduit en morceaux. Quelle erreur ! Les objectifs de santé publique et les intérêts sur le plan économique convergent vers une intégration de l'AME dans le régime général de l'assurance maladie.

une vision d'ensemble, un cap clair. Certaines trajectoires, comme les évolutions de l'AME, mériteraient d'être encore plus affirmées ; d'autres, telle la politique de prévention, ne répondent pas, à ce jour, à nos inquiétudes.

Madame la présidente, madame la ministre, madame, monsieur les rapporteurs, mes chers collègues, le 19 septembre dernier, le Président de la République rappelait que notre système de santé constitue un pilier de notre République sociale et qu'il est l'une des meilleures concrétisations de la solidarité nationale. La mission « Santé » s'inscrit dans cette volonté d'assurer un égal accès aux soins à l'ensemble de nos concitoyens et de corriger les inégalités. Pour autant, si les crédits augmentent globalement de 3,4 %, je regrette que les moyens alloués au programme « Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins diminuent d'un peu moins de 6 millions d'euros. Certains me rétorqueront que c'est bien peu. Certes. Toutefois, comme l'avait souligné le Premier ministre lors de la présentation du plan « Priorité Prévention on meurt trop souvent trop jeune en France. Et une vraie politique de prévention permettrait de préserver près de 100 000 vies par an. » La prévention doit rester au coeur de notre politique de santé. Aussi regrettons-nous, notamment, que les dépenses dédiées à la prévention des addictions connaissent une baisse de 13 %. La France est l'un des pays européens où les adolescents consomment le plus de produits stupéfiants 80 % d'entre eux expérimentent plusieurs produits- tabac, alcool et cannabis -, selon les derniers chiffres de l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies. En revanche, je note avec satisfaction l'augmentation des crédits destinés à soutenir les actions en matière de lutte contre les infections par le VIH, les infections qui passent notamment par le renforcement du dépistage. Selon le dernier bilan épidémiologique publié par Santé publique France, en 2017-2018, 28 % des personnes diagnostiquées pour une infection ont découvert leur séropositivité à un stade avancé et 49 % n'avaient jamais été testées auparavant. Ces chiffres soulignent l'importance du dépistage. S'agissant de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, l'ANSM, je ne peux que souscrire aux propos de notre rapporteure pour avis. J'ai eu l'occasion de le rappeler lors du conseil d'administration de l'agence, la semaine dernière, il n'est pas certain que le maintien de la dotation de l'État à son niveau actuel permette à l'agence de faire face à ses nombreuses missions. Au-delà des missions déjà renforcées depuis 2016, le Sénat a formulé des demandes pour que l'agence investisse les champs suivants l'accès rapide et sécurisé aux innovations thérapeutiques, la prévention et la gestion des ruptures d'approvisionnement de médicaments, son positionnement sur la recherche clinique. Même si je reconnais que l'agence conserve une dotation identique à celle de 2018,

Ma dernière observation porte sur l'AME, qui concentre 99 % des moyens alloués au programme « Protection maladie », avec 935 millions d'euros. Cette année encore, la commission des finances nous demande de diminuer les crédits de l'AME de 300 millions d'euros. Cette proposition ne nous semble pas aller dans le bon sens, et ce pour plusieurs raisons. L'AME se caractérise par une prévisibilité particulièrement complexe, dont découle une sous-budgétisation récurrente. Notre rapporteure pour avis l'a rappelé, réduire cette dépense n'est pas une solution satisfaisante : il faudra la prendre en charge d'une façon ou d'une autre.

L'AME, enfin, constitue une nécessité de santé publique pour éviter la propagation de maladies contagieuses. La commission des finances nous propose également d'instaurer une franchise, comme cela existait avant 2012, pour réduire les dépenses et contrer des abus. Je rappellerai simplement qu'un rapport des inspections générales des affaires sociales et des finances avait jugé une telle mesure financièrement inadaptée, administrativement complexe et porteuse de risques sanitaires.

Madame la présidente, madame la ministre, madame, monsieur les rapporteurs, mes chers collègues,

prévenir les situations à risques et accompagner les personnes pour éviter que les situations ne se reproduisent. Je salue le cap choisi. Nous ne pouvons pas répondre aux enjeux de vieillissement de la population et de développement des maladies chroniques en gardant comme modèle le « tout-curatif La France peut être fière de son système de santé, qui nous permet de jouir d'une des meilleures espérances de vie au monde : 79,5 ans pour les hommes et 85,4 ans pour les femmes.

Nous pouvons en conclure que, si nous vivons plus longtemps, nous vivons aussi longtemps en mauvaise santé, notamment à partir du départ à la retraite. C'est d'autant plus vrai pour les femmes, qui vivent plus longtemps que les hommes, mais ne vivent pas, proportionnellement, plus longtemps en bonne santé. Aussi, la prévention est plus que jamais une urgence pour améliorer les conditions de vie de nos concitoyens, mais aussi pour préserver nos dépenses publiques. Cette ambition portée par Mme la ministre se retrouve-t-elle, par conséquent, dans la mission « Santé » du projet de loi de finances qui nous est présentée aujourd'hui ? La mission « Santé », c'est 1,4 milliard d'euros de budget, réparti entre deux programmes : le programme 204 relatif à la prévention, la sécurité sanitaire et l'offre de soins, pour un tiers de l'enveloppe, et le programme 183 relatif à la protection maladie, qui récolte les deux tiers restants. Si les crédits de la mission progressent globalement de 3,4 %, c'est exclusivement le fait de l'augmentation des moyens de l'aide médicale de l'État, dans le programme 183. À périmètre constant, les crédits du programme 204 diminuent même de 1 %. Aussi, la politique de prévention de la santé devra composer avec 5,5 millions d'euros de moins que l'année passée, comme l'ont déjà relevé un certain nombre d'orateurs. Si la prévention est autant, voire davantage, affaire de changements de pratiques et de mentalité que de moyens financiers, une telle évolution peut être néanmoins regrettée. évolution positive à noter : l'augmentation de plus de 2 millions d'euros des subventions versées à l'Agence nationale de santé publique, acteur majeur de la prévention. Inversement, les sommes versées à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé se réduisent de 120 000 euros, après une augmentation salutaire l'année dernière. Je regrette que le Gouvernement ne maintienne pas l'effort,

Face à la pluralité de ses missions, il convient de donner à cette agence les moyens adéquats. J'en viens maintenant au programme 183, « Protection maladie », qui concentre ses crédits sur l'aide médicale de l'État, Aussi certain qu'après le jour vient la nuit l'AME fait l'objet d'un débat animé à chaque projet de loi de finances. Il serait donc tentant de reprendre, à ce stade, les éléments de l'intervention que j'ai tenue l'an dernier, mais ce serait faire injure à notre assemblée, à nos concitoyens et au débat démocratique. Je tiens à féliciter notre rapporteure pour avis, Corinne Imbert, pour sa prise de position digne et responsable sur le sujet, à laquelle je me rallie bien volontiers. L'AME est une nécessité humanitaire, sanitaire et économique. À sa manière, elle participe à la politique publique de prévention sanitaire.

Mais il serait vain de nous enfermer dans une forme de déni. Les propositions de notre rapporteur spécial, Alain Joyandet, de réduire de 300 millions d'euros les crédits de l'AME et l'instauration d'un droit de timbre annuel pour accéder à cette aide ne me paraissent pas opportunes. Ce droit de timbre tendrait à créer une barrière dans l'accès aux soins, tandis que la menace de réduction des crédits affectés à l'AME n'est plus crédible. Sur ces points, les analyses diffèrent au sein du groupe centriste, je le regrette. Je salue, enfin, la gestion de l'AME de droit commun par les caisses primaires d'assurance maladie de Paris, Bobigny et Marseille. Cet effort de mutualisation permettra des économies de gestion, mais également un renforcement du pilotage du dispositif et du contrôle des dossiers, tout en homogénéisant leur traitement. Pour conclure, si, dans l'intention, le Gouvernement a fait de la prévention son mot d'ordre en matière de politique sanitaire et sociale, d'un point de vue budgétaire, les moyens restent un peu limités. Ces quelques déceptions exprimées, le groupe Union Centriste votera les crédits de la mission « Santé

une dilution du fonds de lutte contre le tabac, élargi, à moyens quasi constants, à l'ensemble des addictions en 2019. La prévention tabac doit être maintenue. Nous saluons, de nouveau, le programme de vaccination mis en oeuvre. Nous saluons aussi la profonde réorganisation du paysage sanitaire présentée par le Gouvernement. La mise en place du Comité d'animation du système d'agences permettra une coordination. Cet effort de cohérence, louable pour renforcer le pilotage des opérateurs sanitaires de l'État, se traduira notamment par une mutualisation des fonctions support. L'ANSM se voit contrainte de repenser son fonctionnement pour faire face au renforcement de ses missions, à la suite de l'entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 2016 de modernisation est attendue face à la multiplication des crises sanitaires, celles du Levothyrox et de la Dépakine, notamment. L'ANSM est aussi mobilisée pour l'accès rapide et sécurisé aux innovations thérapeutiques et pour la prévention et la gestion des ruptures d'approvisionnement de médicaments. Elle est amenée à gérer les conséquences sanitaires du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne. Son budget a été augmenté de 6 millions d'euros en 2018, puis stabilisé en 2019, avec une enveloppe globale de 118 millions d'euros. Sa mission est capitale, notamment pour les ruptures d'approvisionnement de médicaments. Pour lutter contre ce phénomène, il serait nécessaire de renforcer son pouvoir de sanction, comme le préconise la mission d'information du Sénat dont notre collègue Jean-Pierre Decool était le rapporteur, en instaurant des pénalités suffisamment dissuasives pour les entreprises pharmaceutiques. S'agissant de Santé publique France, chargée de la veille sanitaire, ses moyens sont consolidés. moyens sont consolidés. L'agence et l'ANSES sont fortement sollicitées pour objectiver l'impact sur la santé des agriculteurs de l'usage des produits phytosanitaires, mais aussi sur d'autres faits inquiétants, notamment les malformations congénitales observées dernièrement

Plusieurs de ces plans de financement sont incomplets. Seulement 4,5 millions d'euros ont été inscrits dans le projet de loi de finances pour 2019 au sein de la mission « Recherche et enseignement supérieur

sous-budgétisée, comme le démontre sa dette envers l'assurance maladie, qui atteignait 50 millions d'euros en 2017. Ces sommes ne tiennent pas compte des frais engagés par les hôpitaux pour soigner en urgence les étrangers en situation irrégulière non éligibles à l'AME.

La gestion de l'AME sera renforcée en 2019, ce qui est une bonne chose, ainsi que la lutte contre la fraude, qui connaît des avancées importantes. Par conséquent, je soutiens Mme le rapporteur

infectieuses, nécessitant une prise en charge rapide. La lutte contre la fraude enregistre des progrès notables et reste, il nous semble, le seul moyen efficace de prévenir les abus. Le groupe Les Indépendants votera favorablement les crédits de cette mission.

Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le président de la commission des affaires sociales, madame la rapporteur pour avis, monsieur le rapporteur spécial, mes chers collègues, je ne reviendrai pas sur les grandes lignes et les équilibres des crédits de la mission « Santé » du projet de loi de finances pour 2019. Mes collègues rapporteurs ont parfaitement souligné le déséquilibre important entre les deux programmes de la mission et les difficultés que rencontrent aujourd'hui les opérateurs, en raison de budgets qui ne sont pas toujours en adéquation avec les exigences imposées. rappelons-le aussi, ne représentent qu'une toute petite partie des moyens de notre politique publique de santé, qui relève plus largement de la loi de financement de la sécurité sociale. Je souhaitais, pour ma part, insister sur la question de la veille et de la sécurité sanitaires. En tant qu'administrateur de Santé publique France, je mesure le champ toujours plus vaste sur lequel l'agence mais aussi l'ANSES sont et seront mobilisées dans les années à venir. On se souvient du rôle central que ces organismes ont joué dans le dossier de l'amiante ; ils travaillent aujourd'hui sur les conséquences de l'utilisation des produits phytosanitaires chez les agriculteurs, mais mènent également des investigations sur les cas de malformations congénitales récemment signalés. Cette semaine encore, Santé publique France mène des investigations en Haute-Savoie sur des cas signalés de toxi-infections alimentaires, liées à une souche particulière de salmonellose. Son expertise, parfaitement indépendante, doit être saluée. Même si leur budget est consolidé cette année, il conviendra d'être vigilant pour conforter les moyens de ces agences de veille sanitaire : on ne peut constater le nombre croissant de leurs saisines et missions et, dans le même temps, leur demander de réduire leur plafond d'emplois de 2,5 Cependant, pour réaliser ses missions, l'agence s'appuie sur des partenaires, acteurs de terrain. L'implication des professionnels de santé dans la veille sanitaire, au travers des signalements qu'ils réalisent, de leur participation à la réponse aux alertes et de leur interface avec l'usager en relais des politiques de santé, est effectivement un des maillons essentiels de la politique de prévention. Je veux ici souligner l'importance du rôle des médecins généralistes, qui sont de véritables sentinelles en matière de veille sanitaire et sont témoins des inégalités sociales de santé, très marquées entre les différentes catégories socio-professionnelles, mais aussi dans nos territoires. C'est bien en permettant à tout un chacun, particulièrement aux publics les plus défavorisés, d'accéder à une offre de soins au plus près de leurs besoins que la politique de prévention sera la plus efficace. Le constat est largement partagé : plusieurs mois d'attente pour consulter un spécialiste, des médecins généralistes débordés qui ne peuvent plus prendre de nouveaux patients, Lutter contre les déserts médicaux est donc une priorité, car la situation risque encore de se dégrader si rien n'est fait. Les zones rurales ne sont pas les seules concernées : les centres des grandes villes, qui présentent un coût d'installation particulièrement élevé pour un jeune médecin, connaissent également une désertification massive.

de cette problématique de désertification médicale, madame la ministre, vous avez proposé des mesures déjà testées pour garder et attirer les médecins- aides à l'installation dans les zones sous-dotées, simplification de l'exercice mixte salariat-libéral, activité des médecins retraités, développement et remboursement des actes de télémédecine -, mais ces mesures n'ont pas toutes été évaluées à ce jour. Qu'en est-il exactement ? Enfin, nous avons bien conscience que les crédits de la mission « Santé » s'inscrivent, plus globalement, dans le cadre de la stratégie nationale de santé lancée à la fin de 2017, mais aussi dans celui, plus ambitieux, du plan « Ma santé 2022 » présenté en septembre dernier. Il nous faudra être vigilants sur ces différents points,

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, en France, nous avons le privilège et la chance- il faut en avoir conscience -d'avoir un système de solidarité comme il en existe rarement dans le monde, protégeant les plus vulnérables par l'effort national. L'État garde aujourd'hui une place essentielle dans la prise en charge des soins des Français. Son rôle régalien est d'assurer une mission de service public auprès des citoyens n'ayant pas accès à l'offre de soins. de soins. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale et la mission « Santé » du projet de loi de finances programment un budget à cet effet. Parmi les dispositions, l'aide médicale de l'État a pour but de soigner les étrangers arrivant en France, dans un souci d'action sociale et humanitaire. C'est essentiel. L'aide médicale pour soins urgents, qui est vitale, est évidemment une nécessité. 95 % du budget de l'AME est consacré aux étrangers en situation irrégulière, la quasi-totalité de ce budget est réservée, non pas aux soins vitaux, mais à l'aide médicale de droit commun, laquelle couvre, à 100 % et sans avance de frais, les soins quotidiens et de confort. Cette dernière a progressé de 11 % depuis 2015, avec un nombre de bénéficiaires en hausse constante. Je voudrais souligner tout de même, en tant qu'élue d'un département rural où la démographie médicale est particulièrement faible, que l'accès aux soins est un luxe pour certains. certains. Je rencontre souvent des personnes qui ne peuvent pas se payer des lunettes ou des soins dentaires, faute de moyens suffisants. Les crédits alloués en 2019 au programme « Protection maladie », dont dépend l'AME, représentent 944 944 millions d'euros, soit deux fois plus que le programme consacré à la prévention, la sécurité sanitaire et l'offre de soins, et 53 millions d'euros de plus par rapport à l'an dernier. Ces crédits ne cessent d'augmenter. les fonds du programme « Protection maladie » connaissent une croissance de 27 % depuis 2013, alors que ceux qui sont consacrés à la prévention ont diminué de 25 % sur la même période. spécial de la commission des finances évoque d'ailleurs un « dynamisme non maîtrisé des dépenses du programme 183 » et de « carences persistantes dans la stratégie de pilotage raison pour laquelle la commission des affaires sociales appelle, dans les plus brefs délais, à la mise en place d'un référentiel d'évaluation et de projection solide de la dépense de l'aide médicale de l'État. le plan général, les crédits de paiement de la mission « Santé » demandés pour 2019 s'élèvent à 1,423 milliard d'euros, soit 3,5 % d'augmentation par rapport à 2018. Il s'agit d'une augmentation de crédits plus faible que les années précédentes, cette faiblesse s'expliquant par la trajectoire pluriannuelle des finances publiques, qui demande un effort financier soutenu, notamment aux opérateurs sanitaires. On peut se réjouir d'une baisse significative de la dette de l'AME, qui passe en dix ans de 246 millions à 49 millions d'euros. On note également une amélioration de la gestion de l'AME, en partie due à l'efficience de la lutte contre la fraude. Soulignons aussi que ces crédits sont inférieurs au plafond inscrit en loi de programmation des finances publiques. Cette démarche de sincérité budgétaire est une heureuse nouvelle, puisque, comme vous le savez, mes chers collègues, les plafonds de crédits avaient été dépassés Sous réserve de l'adoption des amendements, je voterai en faveur des crédits de la mission. Mes chers